Madame la présidente-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

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des salles de réunion et des circulations du Sénat. Il vous est donc demandé de bien vouloir en porter un dans l'hémicycle.

mais nous avons une faculté de travailler ensemble. Je pense que c'est très bien pour notre République. Merci,

qui sont formés. Je les partage d'autant plus que je suis dans la même situation que vous : il s'agit de ma dernière séance, et de ma dernière prise de parole dans l'hémicycle. Voilà une quarantaine d'années que je suis dans la vie publique et je comprends

qui n'est pas seulement officiel, mais qui est aussi amical, et que je voudrais particulièrement chaleureux. La personnalité très

l'engagement dont vous avez fait preuve dans vos fonctions, tant pour représenter votre territoire, auquel vous êtes tellement attachée que vous souhaitez désormais ne plus le quitter, que comme législatrice. J'ai le souvenir de nombreux textes que vous avez rapportés à la commission des lois, dont vous avez été la vice-présidente. Je pense à celui sur les

Madame la présidente, qu'il me soit permis à mon tour de vous souhaiter bon vent, des alizés peut-être au goût sucré ... Vous avez présidé mes premières séances remercie de votre attention bienveillante. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de défendre aujourd'hui devant votre Haute Assemblée un projet de loi organique

au lendemain de ma nomination. C'est donc un privilège de le soumettre ce matin à votre examen. Surtout, ce texte marque la traduction concrète de la volonté du Président de la République de répondre à une aspiration apparue entre 2017 et 2019, mais qui couvait en réalité depuis bien plus longtemps bien plus longtemps : celle d'un changement de la vie politique pour laisser davantage de possibilités d'expression et d'action à des personnes qui en sont habituellement éloignées, afin de mieux la transformer. transformer. Mais ce changement ardemment désiré est aussi et avant tout celui d'un renouveau de nos institutions et de leur fonctionnement. nos concitoyens ont appelé de leurs voeux une mutation des pratiques politiques, en particulier de notre démocratie représentative. C'est pourquoi, pour répondre à cette attente légitime, le Président de la République a proposé aux Français de moderniser notre démocratie en rendant nos institutions plus représentatives, plus responsables et plus efficaces. Le projet de réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui vous sera présenté à l'automne en sera la traduction concrète. Ce sera, je l'espère, un grand moment de débat démocratique,

Il s'agira, notamment, de permettre au CESE d'organiser des conventions citoyennes, sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, en tirant des citoyens au sort pour organiser une consultation sur un sujet, afin que cet organe devienne la chambre des conventions citoyennes, de renforcer l'importance de ses avis dans le processus législatif et de voir sa composition modifiée pour renouer avec sa vocation initiale de représentation de la société civile. Ce n'est toutefois pas ce texte que je vous présente aujourd'hui. En effet, pour nous permettre d'avoir cette discussion si nécessaire sur nos institutions et leur fonctionnement dans un temps long, propice au consensus et à la coconstruction,

du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, ce mandat a débuté le 15 novembre 2015 et doit s'achever au mois de novembre 2020.

présent projet de loi organique, qui se compose d'un article unique, vise à prolonger le mandat des membres du Conseil pour la durée strictement nécessaire à l'adoption de la loi organique modifiant la composition et aux opérations de renouvellement consécutives à sa publication. Une date butoir est néanmoins prévue, afin que la prorogation du mandat ne puisse pas excéder le 1 juin 2021. C'est pourquoi je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d'adopter le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres actuels du Conseil économique, social et environnemental. La parole

lois au cours de ces dernières années. Le Conseil économique, social et environnemental est la troisième assemblée constitutionnelle de la République. Il a vocation à représenter la société civile organisée.

été pris, du fait notamment de la crise sanitaire et des processus préalables à la nomination des représentants d'un certain nombre de corps constitués, la commission des lois propose d'accepter le projet de loi organique qui nous est soumis. Toutefois, cela ne préjuge en rien

et de garantir le contrôle par des élus de l'ensemble de l'administration d'un État. Il est donc absolument indispensable que la démocratie représentative puisse continuer à vivre. Les débats sur le tirage au sort

Pour autant, et je souhaite le réaffirmer ici, le vote formulé aujourd'hui ne constitue en aucune manière un accord sur l'ensemble de la réforme qui nous est proposée. Nous devrons prendre le temps du débat sur le rôle du CESE et son utilité à l'automne,

à la qualité de la loi du fait de la représentation spécifique des territoires. Dans le détail de la réforme présentée, trois problématiques nous semblent majeures.

qui consistent à abattre un maximum de travail en un temps record, limitant drastiquement le débat et la pluralité des échanges. Ensuite, nous pensons qu'il faudra avoir un vrai débat sur les modalités de participation citoyenne, notamment la place du tirage au sort. La question a été largement ouverte par la Convention citoyenne pour le climat. Si le tirage au sort peut se justifier ponctuellement, cette procédure interroge sur les légitimités ainsi créées et les stratégies

Nous prônons, plus positivement, non pas la création d'un espace concurrent, mais bien le renforcement des possibilités de coconstruction, d'échanges et de débats propices à l'expression de cette parole spécifique. Encore faut-il que le Gouvernement la prenne en compte, bien

Sur le fond, le devoir d'innovation démocratique qui nous incombe, notamment au regard du taux d'abstention constaté aux élections, dépasse les formes d'expression citoyenne pour toucher aux modalités concrètes de partage des pouvoirs et de représentativité de nos institutions. Enfin, nous sommes extrêmement

proposée par le Gouvernement pourrait supprimer certaines compétences dévolues à des organismes consultatifs, et donc potentiellement porter atteinte à la démocratie sociale. Le Conseil d'État lui-même déplore, dans son avis, une mauvaise appréciation du champ d'application de cette mesure. Au fond, nous devrons, lors de nos prochains débats, rendre plus nettes les motivations profondes du Gouvernement, qui pourrait voir dans cette réforme une occasion de discréditer la représentation des corps intermédiaires, sous couvert

chargé, dès sa création en 1925, de représenter les forces économiques et sociales du pays. Sa composition et ses attributions n'ont cessé d'évoluer, s'adaptant aux besoins de la société civile. Il comprend aujourd'hui 233 membres- l'effectif maximal

qui a été déposé le 7 juillet dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je me réjouis que la commission des lois ait admis la prolongation du mandat des membres du CESE, car s'y opposer aurait eu pour effet de renoncer à la possibilité même de réformer

concilier l'affirmation du tirage au sort et la légitimité des urnes, fondement même de notre pacte républicain ? La réduction de 25 % des effectifs du CESE se justifie-t-elle vraiment ? Quelles en seraient les conséquences sur la représentation de la société organisée ? Peut-on renvoyer à un décret la liste des organisations représentées dans les pôles « cohésion sociale » et « protection de l'environnement », alors qu'elle figure aujourd'hui dans la loi organique ? Comme l'a justement souligné l'excellent rapporteur, pour pouvoir débattre de tous ces sujets, vraisemblablement au cours de l'automne, il nous faut dès à présent proroger le mandat des membres actuels du CESE.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 29 juin dernier, le Président de la République a témoigné de sa volonté de transformer le CESE en ce qu'il a nommé la « chambre des conventions citoyennes

le rôle du CESE dans le développement de la démocratie participative. Car, s'il est en effet un acteur essentiel de la démocratie sociale, par sa culture du consensus, dans un pays où les conflits sociaux sont légion, il peine toujours, après tant d'années d'existence, à trouver sa place dans les institutions. Ses travaux, pourtant nombreux et rarement lacunaires, souffrent d'un grand manque de visibilité. Sans surprise, ils sont peu connus du grand public, ce qui s'explique facilement par le manque de lisibilité des nombreux organismes consultatifs qu'abrite la France. également loin, parfois, de l'attention des pouvoirs publics, ce qui est plus inattendu. La concurrence des nombreux autres organes consultatifs en est très probablement l'explication la plus plausible. Pire encore, l'institution du dialogue social est très peu sollicitée, 79 % de ses travaux résultant d'une autosollicitation. Cette institution, troisième chambre prévue par notre Constitution, mérite donc une réforme qui lui attribuerait la place qui lui revient au sein de la République. Celle-ci interviendra au début de l'année 2021, ce qui nous pousse à prolonger le mandat des 233 membres du Conseil, supposé expirer le 14 novembre 2020 après cinq ans de loyaux services. Cette prorogation doit bien évidemment courir jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite réforme. Cependant, si nous convenons de la nécessité d'une réforme, la teneur exacte de celle-ci suscite débat. Assurer un meilleur fonctionnement du CESE pour mieux faire participer les corps intermédiaires au débat public ? Nous partageons tous cet objectif. Veiller à ce que les travaux du CESE reçoivent les échos qui leur sont dus ? Cela va de soi. Doter le CESE des outils dont il a besoin pour accomplir ses missions ? Nous ne pouvons pas nous y opposer. Toutefois, à la lecture du texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, nous nous interrogeons déjà sur certains points. La première réserve concerne le rôle de représentation de la société organisée la réduction de ses effectifs de 25 %, qui porterait le nombre de ses membres à 175, pourrait être lourde de conséquences pour cette noble tâche. autre aspect de la réforme suscite d'ores et déjà le scepticisme, le recours au tirage au sort, qui, jour après jour, prend une place de plus en plus importante dans certains esprits. Si beaucoup chantent les louanges d'un modèle démocratique athénien, le tirage au sort n'en reste pas moins en contradiction totale avec le principe de démocratie représentative si cher à la majorité de nos concitoyens, et qui constitue l'un des fondements de notre histoire politique. chers collègues, méfions-nous de cette douce chanson qui fait l'éloge de la démocratie participative et directe, devenue depuis peu le fer de lance du dégagisme et du populisme. Méfions-nous du tirage au sort, non pas en raison d'une quelconque crainte de nous voir concurrencés dans notre rôle de représentation nationale, mais parce qu'il est tout aussi attirant que dangereux pour les fondements de notre pacte républicain. La place qui est réservée au tirage au sort dans ce projet, nous en conviendrons, n'est pas scandaleuse en soi. Mais cette réforme consacre tout de même le tirage au sort dans la loi, promettant ainsi un avenir institutionnel à cette pratique. Il faut y penser.

Dans l'immédiat, et justement pour que ce débat de fond puisse avoir lieu sereinement, nous voterons en faveur de la prorogation du mandat des membres du CESE prévue par le présent projet de loi organique. La parole est à Mme Christine Lavarde.

À cette heure, et sans préjuger des débats ni du contenu du texte qui nous sera transmis par les députés, je rappelle l'attachement du groupe Les Républicains au rôle que la Constitution accorde à chaque chambre et chaque institution. C'est vrai pour le CESE comme pour le Sénat. Le CESE est un acteur important de la démocratie sociale depuis près d'un siècle. Son rôle a été reconnu en 1958 et il participe depuis lors à l'équilibre constitutionnel.

ce projet de loi vise à reporter le renouvellement des membres du CESE au 1 juin 2021, dans l'attente d'une réforme qui serait destinée à lui donner un nouveau souffle et une nouvelle visibilité, non seulement comme l'enceinte de la représentation des acteurs de la société civile, mais aussi comme un véritable carrefour de la consultation publique et de la participation directe des citoyens. Sur le plan du calendrier, il n'y a pas de débat, la prorogation du mandat de ses membres est indispensable à l'examen préalable de la réforme envisagée. Toutefois, l'adoption de ce texte ne doit en rien présager de la position du Parlement, en particulier du Sénat, sur le projet de loi organique réformant le CESE. Sur le texte examiné ce matin, mon propos pourrait s'arrêter là. Mais son examen en commission des lois a fait l'objet de différentes appréciations, et les pistes d'évolution du rôle et des méthodes de l'institution ont été largement évoquées. Avant d'envisager de nouvelles orientations, il conviendrait de faire un diagnostic de l'activité du CESE au cours de ces dernières années, voire de ces dernières décennies. Sans revenir aux objectifs qui lui étaient fixés dans la Constitution de la V République, rappelons, comme l'indique le rapport de la commission, que le CESE devrait remplir trois missions principales : conseiller le Gouvernement sur les politiques économiques, sociales et environnementales, favoriser le dialogue entre les forces vives de la Nation et contribuer à l'information du Parlement.

l'expression d'une grande autonomie, mais surtout la preuve du peu d'intérêt qui est réservé à ses travaux. Faut-il de surcroît remarquer que les 20 % de saisine par le Gouvernement relèvent d'une démarche obligatoire pour les lois à caractère économique, social ou environnemental On peut aussi noter que le CESE, pour l'étude de certains sujets, est concurrencé par de nombreux autres organismes consultatifs plus spécialisés, et donc mieux outillés pour aborder en profondeur certaines thématiques. Ces doubles emplois emplois risquent encore de s'étendre, notamment à travers la concurrence qui ne manquera pas de s'installer avec la Commission nationale du débat public dans un rôle d'organisateur de la participation directe des citoyens et de la consultation publique. Par ailleurs, il faut noter que la saisine par voie de pétition sur toutes les questions à caractère économique, social et environnemental, possible depuis 2010, n'a jamais été mise en oeuvre. Le CESE ne joue pratiquement aucun rôle opérationnel dans la consultation des corps intermédiaires, qui préfèrent s'adresser directement au Gouvernement et au Parlement pour faire valoir leurs avis et préoccupations. Je n'évoquerai pas la déclinaison régionale du CESE que sont les CESER, dont l'apport réel dans l'élaboration des politiques régionales est tout à fait illusoire ou marginal. À l'occasion de l'examen de la loi NOTRe, j'avais d'ailleurs déposé des amendements visant à supprimer ces instances. instances. Sans remettre en cause son indépendance, la qualité de ses membres ou la pertinence de certains de ses avis, il convient, au vu de ce diagnostic, de s'interroger sur l'utilité du CESE. Cette prolongation du mandat de ses membres permettra quand même de donner une chance à la réforme envisagée, et même souhaitée, par le Président de la République. Elle donnera sans doute lieu dans cette enceinte à des débats animés, qui pourraient qui pourraient entre autres révéler un goût très modéré du Sénat pour la démocratie du tirage au sort. Dans cette attente, le groupe du RDSE approuve le texte de prorogation qui nous est proposé. La parole

le projet de loi organique qui nous rassemble aujourd'hui, nonobstant son caractère formel, n'est pas un texte mineur. Aux termes de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, le mandat de ses membres, d'une durée de cinq ans, arrivera à échéance le 14 novembre prochain. Or, le 7 juillet dernier a été présenté en conseil des ministres un projet de loi organique réformant le CESE. Ce texte prévoit notamment, en son dernier article, que ses dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. Le calendrier ne permettra pas que cette réforme puisse être adoptée et promulguée, à l'issue d'un débat approfondi puis d'une décision du Conseil constitutionnel, avant l'expiration du mandat des membres actuels du CESE. Le Conseil d'État a, en outre, souligné dans son avis la nécessité que le Gouvernement prépare les décrets d'application concomitamment aux travaux parlementaires sur cette réforme, ce qui implique un enjeu de temporalité qui ne peut être éludé. Toutes ces raisons ont conduit le Gouvernement à soumettre à nos voix le présent texte, qui vise donc à proroger le mandat des membres du CESE jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi organique réformant cette

Comme le souligne l'avis du Conseil d'État, une telle prorogation ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel ni conventionnel. Une précédente prorogation avait d'ailleurs été validée dans le cadre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, pour une durée qui était supérieure. Cette simplicité apparente du dispositif appelait en réalité une certaine approche de la Haute Assemblée, et plus spécifiquement de notre rapporteur, la raison d'être du texte étant directement liée à la perspective de l'examen ultérieur d'un projet de réforme. Refuser le principe d'une prorogation aurait conduit à s'opposer à la tenue d'un débat sur la réforme du CESE., accepter cette prorogation était irréductible irréductible à l'expression d'une position sur le contenu de la réforme. Cela ne préjuge en rien du positionnement sur le fond, certes, mais témoigne en revanche- je voudrais saluer sur ce point notre rapporteur, Jean-Yves Leconte -d'une volonté que puisse se tenir un débat sur l'évolution de cette assemblée consultative animée par la culture du consensus, qui ne peut être négligée. L'existence même de cette réflexion, au-delà du contenu du projet de réforme, est invoquée depuis un temps certain, non seulement par le Président de la République et par le Gouvernement, mais également par le CESE lui-même. La part croissante et paradoxale des autosaisines, qui devrait atteindre 80 % en 2020, nous y invite en tout cas, de même que la nécessité de réaffirmer la place de cet organe consultatif dans les institutions, face, tantôt à la défiance, tantôt à l'insuffisante connaissance dont elle peut faire l'objet aujourd'hui. Je salue donc l'adoption par notre commission des lois, sur proposition de notre rapporteur, du présent texte de prorogation. Je veux également saluer la la coordination à laquelle il a procédé, formelle certes, mais qui fait pleinement sens et ne pouvait pas ne pas être, notamment au regard du rôle récent de l'institution dans l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat. présenté tout à l'heure une clarification rédactionnelle qui paraît bienvenue. En conclusion, mes chers collègues, je n'allongerai pas plus mon intervention en m'attardant sur le contenu de la réforme,

pour reprendre la formule si juste de Montaigne, afin de trouver ensemble les modalités d'une juste conciliation entre les différentes expressions de la démocratie et de l'aspiration à la chose publique. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

qui m'offre dix minutes de temps de parole, alors qu'une seule serait déjà de trop pour dire qu'il est inutile de répéter ce que tous les collègues ont excellemment exprimé, à savoir qu'il est judicieux de proroger d'un an le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental ! Je pourrais en rester là, mais ce serait tout de même désobligeant pour notre institution, qui a bien voulu me gratifier des neuf minutes qui restent.

poursuivre la réflexion et être parfaitement au point à la rentrée. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il s'agissait du premier texte que vous souteniez devant le conseil des ministres. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire ...

Lorsque le Gouvernement décidera de consulter le Conseil économique, social et environnemental sur un projet portant sur les questions économiques, sociales et environnementales, le Gouvernement ne procédera pas

consiste à choisir des hommes et des femmes qui défendent des positions et s'engagent sur des programmes et des projets. Il est

publication soit en réalité diffusée sur un site internet que personne ne regarde. Par conséquent, la loi perd de son sens. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi

que le Conseil économique, social et environnemental soit constitué de représentants effectifs des différentes forces économiques, sociales et environnementales

associées relève du champ réglementaire et pourra être réglée par décret simple. Tout à fait ! S'agissant du tirage au sort, il vous vient à l'esprit le sondage, il me vient à l'esprit la cour d'assises,

que vous vous êtes emparé de ce texte, que je me suis contenté de lire et dont je ne suis pas, vous l'avez souligné avec beaucoup d'honnêteté, le rédacteur.

M. le président de la commission. Je voudrais d'abord apporter mon témoignage en faveur du Conseil économique et social devenu Conseil économique, social et environnemental. tant que parlementaire et, dans une vie antérieure, au service de l'État, j'ai observé à de nombreuses reprises la qualité

ces organisations s'opposent. C'est dire que je crois que le général de Gaulle, quand il a souhaité la création de cette institution, a bien fait de vouloir que, à côté du Parlement, qui seul représente la Nation dans sa diversité, il y ait non pas une chambre ou une assemblée, mais un conseil qui puisse être le réceptacle de l'expression de ce qu'on appelle dans notre pays ce n'est pas parce que l'on est reconnaissant au Conseil économique, social et environnemental de son travail au service du pays que l'on doit se laisser entraîner vers des dérives qui seraient, je dois le dire, assez toxiques pour le respect des valeurs fondamentales de la démocratie. Je souhaite

une instance consultative qui permet de prendre en compte les points de vue divers de ceux qui représentent l'économie et la société. C'est un rôle important, mais le Conseil économique, social et environnemental doit rester à sa place s'il veut que sa légitimité soit pleinement assurée. Cette légitimité ne saurait être concurrente de celle de la représentation nationale, mais seulement complémentaire. J'espère que, sur ce point, le Gouvernement et nous pourrons converger, il me semble qu'il existe un risque de dévalorisation de nos institutions démocratiques lorsque l'on prétend qu'il y aurait dans notre pays trois assemblées représentatives, dont les présidents à égalité de dignité pourraient être une sorte de collectif

la qualité démocratique que l'on prête à cet instrument curieux qu'est le tirage au sort. En ce qui me concerne, je n'ai pas suffisamment d'imagination pour considérer que le tirage au sort aurait une quelconque supériorité par rapport à l'expression du suffrage universel. Si ce que je dis est le produit d'une idéologie conservatrice, voire réactionnaire, il faut m'en informer immédiatement ! Elle peut-être, en déformant la réalité historique, tant et tant admiré ceux qui se sont battus pour permettre à nos pères, puis à nos mères de s'exprimer par le suffrage universel pour former cette volonté générale que le Parlement doit incarner que j'ai vraiment du mal à mettre à jour mes conceptions démocratiques et que je n'arrive pas à entrevoir la valeur démocratique du tirage au sort. Qui plus est, le tirage au sort que l'on a mis en oeuvre à travers ce qu'on a appelé de manière si prétentieuse la Convention citoyenne n'est pas un tirage au sort n'est pas un tirage au sort dont les effets seraient naturels. Premièrement, parce que l'on a mêlé au tirage au sort les techniques

Deuxièmement, parce que les personnes tirées au sort se sont, dans leur écrasante majorité, récusées, ce qui fait que, en quelque sorte- pardonnez-moi cette expression triviale -, il n'y a que le fond du panier

il faut tout de même rappeler que les personnes tirées au sort- 150 sur 66 millions d'habitants -représentent 1/440 000 de la population française et n'ont reçu aucun mandat de personne. Par conséquent, il n'est pas démocratique, disons-le haut et fort, de postuler par avance que le fruit de leurs travaux devrait être repris par l'exécutif ou le Parlement ou soumis au suffrage universel par la voie du référendum pour une sorte de validation par oui ou par non sans délibération.

Si nous votions contre ce texte qui prolonge le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental et que le Parlement décidait de diminuer le nombre de membres de cette institution, cette diminution

de la VRépublique ont eu pour seuls objectifs de recaser des battus du suffrage universel ou de faire plaisir à tel ou tel proche du pouvoir.

de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Le scrutin est ouvert.

Madame la présidente,